L'Élysée a indiqué que les deux dirigeants partagent « la même volonté de voir se former un gouvernement crédible » au Liban pour sortir ce pays de la crise, et jugent que sa formation « reste la condition à la mobilisation d'une aide internationale à plus long terme le mois d'octobre dernier, les échanges entre le Premier ministre Saad Hariri et le Président Michel Aoun n'ont toujours pas permis de former un gouvernement, alors que le Liban traverse une crise économique très grave : chute de la livre libanaise, hyperinflation, explosion de la pauvreté, défaillances dans le système de santé et risque de panne énergétique généralisée. C'est cette faillite de l'État qui avait alimenté les manifestations du peuple, lequel réclamait le départ de toute la classe politique et le refus des ingérences étrangères, en particulier iraniennes. Le système politique est empêtré dans ses querelles confessionnelles et la corruption, et reste complètement dépassé par la crise économique. En outre, les résultats de l'enquête sur les causes de l'explosion se font attendre, et il est difficile pour la justice libanaise de travailler en toute transparence, à l'abri des interférences politiques. Lors de son dernier déplacement à Beyrouth, en septembre dernier, le Président de la République avait posé la formation d'un gouvernement légitime comme condition à la mobilisation de l'aide internationale, en particulier dans le cadre des conférences Cèdre en lien avec la Banque mondiale. L'heure n'est-elle pas venue de faire preuve de plus de fermeté pour y parvenir et, ainsi, porter urgemment une aide secourable et nécessaire à la population libanaise ? comment comptez-vous renforcer la pression de la communauté internationale, en particulier de l'Union européenne, pour soutenir le peuple libanais ?

Cette crise n'est pas liée à une catastrophe naturelle : elle a des responsables bien identifiés. Face à cette situation, les forces politiques libanaises refusent de s'entendre sur la composition d'un gouvernement : leur aveuglement est un crime de non-assistance à pays en danger. Pourtant, vous l'avez rappelé, des engagements avaient été pris le 1 septembre dernier, y compris sur la totalité des réformes à entreprendre, que chacun connaît. L'obstruction délibérée à toute perspective de sortie de crise, en particulier de la part de certains acteurs du système politique libanais, par des demandes inconsidérées et d'un autre temps, doit cesser Je vous informe, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que des propositions concrètes sont en cours d'élaboration à l'encontre de ceux-là mêmes qui ont abandonné l'intérêt général au profit de leurs intérêts personnels. Si certains acteurs politiques libanais ne prennent pas leurs responsabilités, nous n'hésiterons pas à prendre les nôtres. Les décisions qu'ils prendront ou qu'ils refuseront de prendre au cours des prochains jours seront déterminantes. est le message que le Président de la République et moi-même avons adressé aux principaux responsables libanais hier. La France, pour sa part, continue de se tenir aux côtés du peuple libanais. Nous savons que le Liban peut compter sur des Libanaises et des Libanais de valeur, au sein de la société civile, qui ont à coeur de travailler sincèrement à l'édification du Liban de demain.

elle ne portera pas sur le sort d'une subvention de 8 000 euros allouée à l'aéroclub du Poitou ou sur le « péril vert » d'une police des rêves d'enfants. Suffisamment de ministres ont surréagi là-dessus, et continueront sans doute à le faire lors des prochains épisodes de la série « Haro sur les écolos ? Ma question porte sur le nécessaire soutien au secteur aéronautique, qui est l'un des plus durement frappés par la crise mondiale provoquée par la pandémie

d'Air France participe de cet effort public. Il serait cependant illusoire de penser qu'il suffit de milliards payés par les contribuables pour assurer un avenir durable à l'aérien secteur ne peut s'exonérer d'une transition qui réponde aux enjeux sociaux, économiques et climatiques. Quelque 400 000 emplois sont en jeu pour l'ensemble du secteur. Nous ne pouvons pas accepter le délitement et les suppressions programmées.

à ce que chacun d'entre nous, pour l'ensemble de son bilan carbone, passe sous les deux tonnes par an d'ici à 2050. Quelle est la stratégie pour la décarbonation du secteur ?

le secteur aérien français figure parmi les plus durement frappés par la crise sanitaire. Dans ce contexte, l'État a su prendre les décisions permettant de garantir la pérennité d'Air France et de Corsair. Je souhaite, pour ma part, appeler votre attention sur la situation d'Air Austral, compagnie française de l'océan Indien basée à La Réunion, qui contribue depuis plus de trente ans au rayonnement des ailes françaises dans la zone sud de l'océan Indien. Depuis le mois de janvier 2020, cette compagnie régionale a subi une chute dramatique de son chiffre d'affaires, de près de 55 %, ainsi qu'une dégradation de ses résultats.

qui fait vivre plus de mille familles à La Réunion. Il est urgent de maintenir les capacités de trésorerie de la compagnie. Un financement d'État de 30 millions d'euros était prévu.

pour la sauvegarde de la pérennité de la compagnie. Par ailleurs, quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger Air Austral des velléités d'Air France ?

De désabusement, car jamais leur profession n'a été aussi incomprise et caricaturée D'inquiétude, car les agriculteurs ne comprennent plus quel chemin on veut leur faire prendre. Avant de trancher, il faut revenir à l'essentiel : en quoi une bonne PAC consiste-t-elle ? une bonne PAC consiste-t-elle ? C'est une politique pour une agriculture souveraine, non dépendante des importations d'autres pays. C'est une politique qui favorise le pouvoir d'achat des citoyens, tout en soutenant le revenu des agriculteurs par des aides du premier pilier. C'est une politique en faveur de notre compétitivité, qui n'abandonne pas notre vocation exportatrice. C'est une politique de solidarité entre filières, notamment par la correction des handicaps naturels extrinsèques à la volonté des hommes. (ICHN) doivent être garanties à l'euro près par le budget national. C'est une politique qui invente l'agriculture de demain, en la faisant évoluer et en respectant le temps long des cultures, sans ajouter de contraintes supplémentaires pour nos agriculteurs. ministre, la politique agricole commune que vous envisagez ne va pas jusqu'au bout. C'est ce qui inquiète les filières. Écoutez donc leurs attentes Plus de transferts entre piliers, c'est plus de distorsions de concurrence entre États membres. En France, le taux doit être tout au plus maintenu à son niveau actuel. Les écorégimes ne doivent pas devenir une usine à gaz : ils doivent répondre à des conditions simples et embrasser un maximum d'agriculteurs.

jours des vagues de froid très importantes un peu partout dans notre pays, lesquelles ont des conséquences dramatiques sur plusieurs de nos filières. Cela renvoie d'ailleurs à une question dont nous avons beaucoup discuté, celle de l'assurance récolte dans le monde agricole.

Hier, depuis leur habitation, ce sont donc 12 millions d'élèves qui ont tenté de se connecter. Malheureusement, deux séries de bugs informatiques les ont privés d'école, du moins temporairement : le bug de « Ma classe à la maison »,

accusation, d'autant que certains ENT sont hébergés par Amazon. Quant au CNED, c'est l'explication d'une cyberattaque par déni de service qui a été avancée, soit exactement la même que celle qui a déjà été subie en mars 2020.

Pourriez-vous nous expliquer les raisons précises de ces bugs et nous rassurer sur le fait qu'elles sont définitivement résolues ? À la suite de l'attaque subie par le CNED l'an passé, quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle ne se reproduise ? L'État a-t-il dialogué avec les collectivités locales pour qu'elles redimensionnent les hébergements des ENT ? Enfin, de nombreux professeurs sont obligés de contourner ces difficultés en recourant à des plateformes, comme celles de Windows ou de Google. Disposez-vous d'un chiffrage précis sur l'étendue du phénomène ? La

vous avez annoncé une nouvelle aide de 4 milliards d'euros et une montée de l'État au capital d'Air France-KLM à hauteur de 29,9 %, qui lui permettra de redevenir le premier actionnaire de la compagnie. Depuis le début de cette crise, notre groupe n'a cessé de plaider pour des prises de participation de l'État dans les grandes entreprises stratégiques. Vous nous avez répondu que cela était impossible. Votre position a manifestement changé, mais vous avez perdu un an. an. Ce soutien à Air France risque de coûter cher en contreparties exigées par la Commission européenne, au détriment des salariés et des usagers. S'agissant des créneaux qu'Air France va devoir céder à ses concurrents, vous vous félicitez de n'avoir à céder que 18 créneaux plutôt que les 24 demandés initialement par la Commission européenne. Mais exiger d'une entreprise en difficulté qu'elle cède des créneaux, même peu fréquentés et même à des compagnies répondant à certaines exigences fiscales et sociales, ce qui n'est pas de l'avis de la Commission européenne,

Cette prise de participation est-elle temporaire dans le but de nationaliser les pertes puis de reprivatiser les profits dès que la situation s'améliorera, en faisant payer l'addition aux salariés, ou s'agit-il d'un engagement pérenne, bénéfique à Air France, à ses salariés et à ses usagers ?

de notre détermination à soutenir cette compagnie aérienne nationale. Il y va de l'indépendance de la France et de notre capacité à peser dans le tourisme mondial. Des contreparties ont certes été exigées, mais je rappelle tout de même que Lufthansa a accepté de céder 48 créneaux en échange du soutien de l'État allemand. Air France

en apportant un soutien de 4 milliards d'euros à Air France et en en devenant le premier actionnaire, l'État réaffirme son engagement aux côtés de la compagnie et de ses salariés. C'est une action nécessaire pour consolider fortement cette entreprise stratégique pour la France. La question du pass sanitaire ou certificat vert doit également être tranchée pour offrir davantage de visibilité au secteur. Nos compagnies aériennes françaises régionales, soutenues par nos collectivités territoriales, souffrent tout autant. C'est le cas d'Air Tahiti Nui, qui a dû mettre en oeuvre un plan d'économies drastique sans bénéficier du chômage partiel, en se séparant de 17 % de ses salariés. La compagnie, vitale pour la Polynésie française, passera difficilement l'année sans une intervention financière de l'État et l'été sera dramatique, si les frontières polynésiennes ne sont pas rouvertes au tourisme, alors que le contexte sanitaire est maîtrisé là-bas, à 16 000 kilomètres de Paris. Monsieur le ministre, alors qu'Air France va être, à juste titre, soutenue massivement, que comptez-vous faire pour accompagner nos compagnies aériennes françaises régionales, tout aussi stratégiques pour l'économie de nos territoires ultramarins, en particulier Air Tahiti Nui ?

à voler et à desservir ses destinations habituelles. Nous avons besoin de trouver d'autres modalités de soutien que celles que nous avons déjà mises en place. C'est pourquoi j'invite Air Tahiti à saisir le CIRI et à discuter avec nous. Nous trouverons des solutions.

Le 11 mars dernier, le Sénat examinait la proposition de loi de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à établir le droit à mourir dans la dignité.

Quelques députés ont déposé 2 300 amendements. Cette obstruction délibérée empêchera vraisemblablement l'Assemblée nationale de se prononcer demain. Et le Gouvernement dans tout cela ? C'est cette question que de nombreux Français se posent et nous posent. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, vous le savez,

précédent plan s'était terminé en 2019 : il fallait le relancer afin de prendre en compte les enjeux du développement de la prise en charge en ville, de mieux répondre à la nécessité d'améliorer la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels et aussi de mieux sensibiliser nos concitoyens à ces questions. Nos concitoyens doivent, par exemple,

le Gouvernement de réfléchir à une loi sur la fin de vie. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, la noblesse de la politique, c'est d'assumer les débats difficiles avec responsabilité et courage.

Vous aviez alors évoqué de prétendues attaques informatiques venues de Russie. On se demande bien quel pirate informatique russe aurait comme objectif de voler les cours de maths de CM1

En 1979, Renault installait ses activités de fonderie fonte et aluminium à Ingrandes, dans la Vienne. En 2019, quarante ans plus tard, après être passées entre les mains de différents groupes et tout en ayant conservé Renault comme principal donneur d'ordre, les deux branches, fonte et aluminium, en grandes difficultés, étaient cédées au groupe GFG Alliance et à sa filiale Liberty. ans d'une mondialisation loin d'être heureuse, car depuis quelques années le Châtelleraudais compte les pertes d'emplois par centaines. Aujourd'hui, en dépit du soutien du Gouvernement à la reprise par GFG et Liberty en 2019, les deux branches courent à nouveau un grand risque de disparition. Côté fonte, si rien n'est fait, ce sont 288 salariés qui seront sans emploi en juin et sans garantie sur leurs indemnités, puisque nous avons appris récemment que Greensill, organisme de financement de GFG, avait fait faillite. Derrière ces sigles et ces grandes manoeuvres de multinationales, il y a, à Ingrandes, des familles dans le désarroi. Côté aluminium, la même menace plane avec un risque de non-paiement des salaires dès le mois prochain.

Si oui, quelles sont les perspectives pour le secteur de la fonderie, qui dépend de grandes entreprises donneuses d'ordre, dont l'État lui-même est actionnaire ?

que les Fonderies du Poitou, dans leur volet aluminium, soient pénalisées par la situation financière du groupe Liberty, auxquelles elles appartiennent depuis plusieurs mois. De manière plus générale et pour vous montrer que nous avons une stratégie, je veux évoquer de la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique, qui a des conséquences sur des milliers d'emplois dans notre pays. Je tiendrai dans les prochaines semaines, au ministère de l'économie et des finances, une réunion avec l'ensemble des acteurs concernés- organisations syndicales et patronales, représentants du secteur industriel, etc. -pour regarder l'avenir des fonderies en France et des milliers de salariés concernés. Les accompagner, les soutenir et assurer la transition, c'est cela avoir une politique industrielle ambitieuse pour la France

retourner sur le terrain au contact des ouvriers, d'une part, et savoir où sont passés les millions du plan garanti par l'État, d'autre part. C'est le seul « en même temps » qui pourrait montrer un témoignage de sympathie envers les ouvriers. La parole est à Mme Patricia Demas, pour le groupe Les Républicains.

santé (DGS), seule une moitié des professionnels de santé a reçu au moins une injection de vaccin anti-covid, alors que l'ensemble des soignants y est éligible. C'est une priorité au regard du rôle qu'ils remplissent dans la bataille sanitaire qui est la nôtre. Pour un soignant, se faire vacciner est conforme à l'éthique de la profession et s'apparente à une obligation pour protéger nos plus fragiles. Ces fondamentaux doivent s'appliquer d'autant plus que la vaccination diminue considérablement les chaînes de transmission du virus. Pour mémoire, les personnels et les étudiants des professions médicales et paramédicales sont d'ores et déjà soumis à une obligation de vaccination qui varie en fonction de leur lieu d'exercice et de la nature de leurs activités. Dans cet esprit et au regard du contexte, le ministre des solidarités et de la santé appelait dernièrement à la vaccination de tous les soignants contre la covid-19, tout comme le Conseil de l'ordre des médecins. Selon l'Académie nationale de médecine, la pandémie que nous vivons a provoqué la crise sanitaire et économique la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale et a entraîné une hausse sans précédent des infections nosocomiales. Le devoir d'exemplarité s'impose. Cette exemplarité agira positivement sur la confiance des Français dans la vaccination, tout en confortant leur reconnaissance envers une corporation qui n'a jamais failli. Alors que les Français sont une nouvelle fois soumis à un confinement, que compte faire le Gouvernement concernant la vaccination insuffisante des soignants, dans un contexte qui s'est lourdement aggravé et où vacciner est notre priorité ?

Monsieur le secrétaire d'État, vous ne répondez pas à ma question et je vous avoue ne pas comprendre votre frilosité. Mon interrogation était pourtant claire et simple : au regard de la pandémie galopante, le Gouvernement compte-t-il s'engager pour rendre la vaccination des soignants obligatoire ?

Le ministère de la justice a adressé aux procureurs deux circulaires les invitant à recueillir avec attention les plaintes des élus et leur demandant de recourir aux sanctions prévues par la loi. Aujourd'hui, le ministère de l'intérieur met à disposition des élus 350 négociateurs

près de Lyon, qui doit aujourd'hui exercer son mandat sous protection policière. Vous l'avez dit, monsieur le garde des sceaux, les agressions contre les élus sont des agressions contre la République et ces agressions minent la République. Faisons très attention à ce que cette peur qui apparaît chez les élus ne commence pas à rendre plus épars les rangs de l'armée des fantassins de la République dont nous avons besoin- ce sont eux qui la font au quotidien et elle leur doit justice ! La parole La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour le groupe Les Républicains. pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le ministre, dans le cadre du plan de sauvegarde d'Air France, qui a déjà perdu plus de 7 milliards d'euros en 2020, vous avez engagé sa recapitalisation par l'État à hauteur de 4 milliards d'euros, moins d'un an après l'octroi de 7 milliards d'euros en prêts d'État ou Je m'en réjouis, car il y va de notre souveraineté nationale et cela entre pleinement dans nos trois objectifs de prise de participation d'État : les entreprises stratégiques pour la souveraineté nationale, celles qui remplissent des missions de service public et enfin les entreprises en difficulté systémique, mais disposant encore d'un modèle valide. Entre Keynes et Schumpeter, cette crise nous rend tous modestes et pragmatiques, mais aussi volontaristes pour reconstruire un souverainisme industriel que nous avons trop longtemps abandonné.

Le contexte exige cette politique industrielle volontariste de l'État. C'est vrai pour nos entreprises publiques, cela l'est aussi pour nos entreprises privées, en particulier les ETI et les PME. C'est pourquoi ma question porte sur le rendez-vous majeur que nous allons avoir avec nos entreprises en sortie de crise. Elle s'inscrit aussi au carrefour de la mobilisation de l'épargne des Français, estimée à 165 milliards d'euros à la fin de 2021, de l'accroissement de la dette des entreprises et des contraintes que connaissent les banques depuis Bâle II. Nous devons préserver la capacité d'investissement des entreprises. Pour cela, nous devons pouvoir, comme vous le faites pour Air France, transformer des PGE en fonds propres ou, pour les plus petites entreprises, en subvention. Les fonds propres constituent la vraie richesse de notre économie. En 2020, nous en avons détruit 50 milliards d'euros sur l'ensemble de notre système productif. Il nous faut impérieusement réalimenter notre appareil productif et concrétiser notre ambition. Quelles réponses, monsieur le ministre, pensez-vous apporter à nos entreprises

Monsieur le sénateur, je partage votre analyse sur la nécessité d'apporter un soutien clair de long terme à nos entreprises, en particulier aux entreprises industrielles.

Ces entreprises doivent savoir que nous continuerons à les soutenir aussi longtemps que cela sera nécessaire. Rien ne serait pire que de retirer brutalement à ces entreprises les aides qui leur ont permis de garder la tête au-dessus de l'eau pendant les mois de crise que nous avons connue et que nous continuons de connaître. Les entreprises qui sont les plus touchées doivent être les plus soutenues ; elles doivent pouvoir continuer à bénéficier de notre soutien- ce sera le cas. D'autres entreprises ont déjà commencé à retrouver des couleurs et veulent investir,

ne pouvons pas nous permettre de dépendre presque intégralement de l'Asie pour des semi-conducteurs qui servent ensuite dans notre industrie automobile, de dépendre des batteries électriques chinoises ou sud-coréennes alors que nous voulons être indépendants. Nous allons donc recréer une indépendance industrielle sur des chaînes de valeur stratégiques telles que les batteries électriques, le, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'hydrogène. Sur toutes ces filières de production, la France veut et va retrouver son indépendance industrielle.

Pourtant, la loi française du 20 juillet 2011 a reconnu la spécificité du volontariat, qu'elle définit comme un engagement citoyen libre qui ne saurait être assimilé à une charge de travail. La transposition et l'application de cet arrêt inquiètent beaucoup, non seulement les sapeurs-pompiers, mais aussi les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. Cette transposition rendrait en effet impossible la conciliation d'un engagement volontaire et d'une activité professionnelle. Elle pourrait ainsi porter gravement atteinte à notre modèle de sécurité civile, fait de la complémentarité entre professionnels et volontaires, dont la force est unanimement reconnue. le ministre de l'intérieur, vous avez initié, en novembre, une demande auprès des directeurs de SDIS qui laisse penser que la France pourrait se diriger vers l'assimilation des volontaires à des travailleurs, et ce de façon abusive et infondée. Vos deux prédécesseurs, M. Collomb au Congrès national des sapeurs-pompiers à Ajaccio et M. Castaner devant le Parlement, avaient affirmé la volonté du Gouvernement de pérenniser et de renforcer le volontariat, dont nous connaissons l'importance fondamentale sur nos territoires. Pouvez-vous nous préciser vos intentions ?

à Mme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les sapeurs-pompiers volontaires belges devaient être, en raison des circonstances d'emploi contraignantes qui leur sont propres, considérés

nombre d'élus. Les échanges dont le Gouvernement français a pris l'initiative avec la Commission européenne nous ont permis de le confirmer formellement, cet arrêt n'implique aucunement que les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires français soient qualifiés de travailleurs. Le Gouvernement est, comme vous, pleinement attaché au statut particulier et au modèle de volontariat français. Chaque cas d'espèce doit être examiné en fonction de ses caractéristiques propres. Cette décision ne remet pas en cause notre modèle du volontariat. Toutefois, il est vrai, ce modèle nous semble devoir être sécurisé, en traitant les situations locales,

particulièrement en cette période de pandémie. Il ne saurait être question pour nous de rester sans agir pour traiter les fragilités juridiques qui peuvent exister. Sur ce dossier sensible, mais structurant pour le modèle français de la sécurité civile, le Gouvernement veut privilégier la concertation, vous l'avez rappelé. Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs généraux de la sécurité civile et de la gestion des crises de lancer une large concertation sur les nécessaires adaptations du modèle actuel de volontariat. Les messages du Gouvernement dont vous faites mention avaient justement pour but de préparer cette concertation. Elle est menée en liaison étroite avec les SDIS,

comme un travail : c'est un engagement citoyen fort ! Ce n'est pas une étude de quelques cas spéciaux que nous vous demandons. L'ensemble des sapeurs-pompiers de France attend l'écriture d'une nouvelle directive spécifique et non une simple dérogation au cas par cas. La France présidera, en janvier prochain, l'Union européenne : voilà une belle occasion de conclure ce dossier

Cela concerne l'acier, le cuivre, le minerai de fer, le zinc, le verre, mais aussi, dans des proportions très importantes, le bois. Aucune matière première n'est épargnée. Le cuivre a augmenté de 28 % depuis un an, le zinc de 22 %. La livraison de bois est devenue extrêmement difficile. Les matériaux deviennent très rares et très chers. Le phénomène s'est répandu au niveau mondial comme une traînée de poudre ; la tension devrait perdurer encore plusieurs mois. Face à ces hausses brutales, il existe un véritable danger pour les entreprises qui se sont engagées sur des bases devenues obsolètes. Bien sûr, monsieur le ministre, le prix des matières premières vous échappe, mais ces entreprises méritent toute votre attention. C'est dès à présent qu'il vous faut activer des leviers pour agir. Devant cette situation exceptionnelle, ne pensez-vous pas que les règles très strictes qui encadrent la commande publique pourraient être temporairement assouplies ? Ne faut-il pas réfléchir pendant cette période si particulière à la possibilité pour le maître d'ouvrage public, de façon systématique, de revoir les conditions initiales du contrat, qu'il s'agisse du prix ou des délais d'exécution ? Ne faudrait-il pas, afin que nos entreprises passent ce nouveau cap, instiller de la souplesse, en permettant plus aisément et plus rapidement l'application des clauses de révision de prix, même lorsque les marchés ont été signés à prix fermes non actualisables ni révisables ? En outre, face au risque de blocage des chantiers dans les semaines à venir, il convient de réactiver les ordonnances qui, au printemps 2020, avaient transitoirement gelé les pénalités de retard des marchés publics et privés. La

l'Asie, mais également aux États-Unis, sous l'impulsion du plan de relance lancé par le Président Biden. Je souhaite que l'Union européenne ne soit pas à la traîne oeuvre le plus rapidement possible son plan de relance afin de renouer avec la croissance et de rester dans la course économique mondiale aux côtés de la Chine et des États-Unis. Je souhaite également que nous réfléchissions de manière plus stratégique à notre indépendance sur un certain nombre de matériaux.

Cette décision, fondée uniquement sur des considérations environnementales, est actée par le projet de loi Climat et résilience sans qu'aucune concertation avec les élus locaux ait eu lieu en amont. Pourtant, cette navette aérienne transporte jusqu'à 550 000 passagers par an. La métropole bordelaise constitue par ailleurs le troisième bassin d'emploi pour l'aéronautique en France et représente près de 35 000 salariés, avec 300 entreprises, dont Dassault ou Thalès. Alors que la région est déjà fortement impactée par la crise, cette suppression risque de remettre en question le choix de localisation et de développement de nombreuses entreprises. entreprises. Dans son avis sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Conseil d'État critique la suppression de la navette Air France entre Bordeaux et Orly. Il souligne que « les conséquences économiques et concurrentielles de l'interdiction sont trop succinctement abordées ». Il vous reproche aussi, monsieur le ministre, de ne pas avoir pris en compte le principe de liberté des transports aériens, qui prévaut dans l'Union européenne. européenne. J'appelle votre attention sur le fait que l'aéroport de Bordeaux s'est doté d'un plan d'orientation stratégique volontariste en termes de lutte contre les nuisances sonores et visant à la neutralité carbone afin de devenir un équipement écoresponsable. la filière aéronautique travaille ardemment à la fabrication d'avions moins polluants dans le cadre du programme européen Clean Sky. Plutôt qu'une suppression totale de cette liaison aérienne, ne serait-il pas possible d'organiser une transition acceptable en maintenant au minimum deux allers-retours quotidiens ?

entre Paris-Orly et Bordeaux, conséquence de l'article 36 actuellement débattu à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Climat et résilience. Cet article, vous y avez fait référence,

Enfin, les lignes concernées bénéficient toutes d'une liaison ferroviaire de qualité. Des aménagements de fréquence à la hausse, dès que la crise sanitaire s'éloignera, nous permettront de retrouver le niveau de desserte habituel. Concernant Bordeaux, j'ai demandé à Mme la préfète de région d'être d'être particulièrement attentive aux besoins locaux, notamment en termes d'accessibilité et de desserte régionale. Les modalités précises de l'application de cet article seront définies par décret. Je souhaite que les élus y soient étroitement associés. La parole

sous la forme de questions-réponses, sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête ; puis, à la demande du groupe Les Indépendants- République et Territoires, un débat, sous la forme d'une discussion générale, sur le thème : « Écriture inclusive : langue d'exclusion ou exclusion par la langue ? Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Par courrier en date du 6 avril, le groupe Les Républicains demande que le débat sur l'avenir institutionnel, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, inscrit à sa demande à l'ordre du jour du mardi 4 mai, soit organisé sous la forme d'une discussion générale et non d'une série de questions-réponses. Y a-t-il des observations ?

la durée de la discussion générale sur les deux textes inscrits à l'ordre du jour de son espace réservé du jeudi 15 avril. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion du 6 avril 2021, un avis favorable- 13 voix pour, aucune voix contre -à la reconduction de M. Jean-Christophe Niel à la direction générale de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable- 9 voix pour, 20 voix contre -à la nomination de M. Philippe Baptiste à la présidence du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales.

voter contre. Acte est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au et figureront dans l'analyse politique des scrutins. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une sécurité globale

sécurité globale préservant les libertés. La commission mixte paritaire (CMP) réunie le 29 mars dernier à l'Assemblée nationale est parvenue à un accord qui préserve la quasi-intégralité des apports du Sénat, dans le souci permanent de mieux protéger nos forces de l'ordre tout en respectant les libertés publiques.

les prérogatives judiciaires des agents de police municipale en leur permettant de constater davantage d'infractions, sous l'autorité du parquet. Le principal point de désaccord entre nos deux chambres portait sur la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des saisies. Nous avons trouvé en CMP une rédaction atteignant un équilibre, conservant le principe des saisies en matière de vente à la sauvette et de consommation de stupéfiants, mais clarifiant leurs conditions de conservation et de destruction, principales raisons de notre réserve. La proposition de loi comprend également plusieurs articles utiles sur la police municipale. Tous les apports du Sénat sur la mutualisation des polices municipales, l'intervention de l'échelle intercommunale, la création de brigades cynophiles ou encore les prérogatives des gardes champêtres ont été préservés. Sur l'ensemble de ces points, nous sommes parvenus à un accord. Il s'agit d'avancées importantes pour nos polices municipales. Nous avons pu préserver les modalités d'évaluation souhaitées notamment par notre collègue Françoise Gatel. S'agissant de l'article 6, supprimé par le Sénat, la CMP a adopté une proposition de rédaction commune qui fait de ce dispositif une simple possibilité

J'en viens au titre relatif aux forces de sécurité intérieure. S'agissant de l'article 24, la rédaction du Sénat a été adoptée sans modification. Je profite de cette occasion pour indiquer que cette rédaction, comme l'a dit notre président

D'abord, elle crée une infraction dont le libellé montre que celle-ci est sans lien avec la diffusion de données. En effet, la provocation à l'identification que vise désormais l'article 24 peut s'opérer sans diffusion de données. Les deux infractions ne visent donc plus la même chose. Soit il y a provocation à l'identification pour les catégories de personnes visées par l'article 24, soit il y a diffusion de données identifiantes sans provocation et c'est l'article 18 de l'autre loi qui s'applique. Nous avons ainsi purgé le vice initial des deux textes concurrents. Je présenterai un amendement rédactionnel visant à bien distinguer les douaniers en opération des forces de l'ordre en opération de police. de police. L'article 23 constituait le principal point de désaccord entre nos deux assemblées. Nous considérions que, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'article posait des questions au regard des principes d'égalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Nous avions donc choisi de centrer le dispositif sur les infractions les plus graves et d'élargir le champ des victimes concernées. La CMP a conservé les principaux points de cette rédaction, tout en réduisant la durée des crédits proposés.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en complément de l'intervention de mon collègue corapporteur Marc-Philippe Daubresse, que je remercie également pour le travail que nous avons accompli ensemble, j'aborderai plus particulièrement

C'est surtout sur la question de la captation et de l'utilisation des images que des divergences subsistaient entre nos deux assemblées. Nous sommes cependant parvenus à les surmonter grâce au travail approfondi mené avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Mme Thourot et M. Fauvergue, que je remercie également. Avant de revenir sur ce point, j'aimerais évoquer en quelques mots les dispositions relatives à la sécurité privée. Le Sénat partageait pleinement la volonté des députés de mieux encadrer ce secteur, ce qui a favorisé l'élaboration d'un compromis. Concernant la sous-traitance, c'est la version adoptée par le Sénat qui a été retenue, même si certains membres de la commission mixte paritaire auraient souhaité imposer des règles plus contraignantes. Il nous a semblé important que la restructuration du secteur ne prive pas les entreprises de sécurité privée de la souplesse dont elles ont besoin pour répondre aux demandes de leurs clients, qui peuvent être amenés à organiser ponctuellement de grands événements, notamment en 2023 et en 2024. S'agissant de l'accès aux métiers de la sécurité privée, le texte qui vous est soumis est proche de celui qui avait été adopté par le Sénat. La durée de séjour exigée des ressortissants étrangers pour obtenir un agrément est cependant portée de trois à cinq ans. Il s'agit d'un point auquel nos collègues députés étaient très attachés, afin de garantir un contrôle effectif des antécédents judiciaires. En ce qui concerne les pouvoirs nouveaux confiés au Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), nous avions une interrogation sur l'opportunité d'introduire une sanction pécuniaire pour les salariés. Un compromis a été trouvé autour d'un montant plus adapté aux capacités financières des personnes visées, qui sont, comme vous le savez, assez mal payées. Enfin, le débat que nous avions souhaité ouvrir sur l'opportunité d'appliquer aux agents de sécurité incendie les règles applicables aux agents de sécurité privée se poursuivra, une demande de rapport que le Gouvernement devra remettre dans un délai de dix-huit Sur les sujets qui touchent à la captation d'images, le Sénat s'est appuyé sur l'avis rendu par la CNIL à la demande du président François-Noël Buffet. Les garanties introduites ont été préservées. Concernant la transmission des images de vidéoprotection à la police, par exemple depuis les halls d'immeubles ou les gares, nous avons trouvé des compromis pour concilier la lutte contre les incivilités avec la nécessaire protection de la vie privée. Pour ce qui est de l'usage de caméras mobiles par les forces de l'ordre, c'est la version du Sénat qui a été retenue : la consultation immédiate des images en intervention sera possible pour certains motifs opérationnels précis, mais leur diffusion directe dans les médias a été écartée, pour éviter tout risque de « bataille médiatique ». S'agissant enfin du recours aux drones, nous avions souhaité le réserver aux circonstances où ils sont réellement utiles, à savoir les infractions graves, les lieux difficiles d'accès ou dangereux. La CMP a maintenu tous les apports du Sénat, notamment l'exigence d'une autorisation préalable, l'élaboration d'une doctrine d'emploi et l'interdiction du recours à la reconnaissance faciale. Sur proposition du Gouvernement, le Sénat, vous vous en souvenez, avait autorisé à titre expérimental l'utilisation des drones par les polices municipales. Nous avions alors fait part de nos interrogations. Nos collègues rapporteurs de l'Assemblée nationale ont, eux aussi, exprimé des réserves. Nous avons finalement décidé d'encadrer encore mieux cette expérimentation. Elle sera soumise à une délibération du conseil municipal et à une autorisation du préfet. Sa durée sera limitée à six mois renouvelables et son évaluation sera renforcée. Pour finir, je signale que la commission mixte paritaire a trouvé un compromis sur la simplification des modalités de contrôles d'alcoolémie au volant, à laquelle nous étions au départ assez réticents, craignant qu'elle n'entraîne une limitation disproportionnée de la liberté d'aller et venir. Nous avons toutefois admis l'utilité d'une telle mesure sous réserve d'un encadrement renforcé. Pour conclure, je tiens à saluer à mon tour le travail constructif mené avec nos collègues députés, qui a permis de dégager un compromis ambitieux tenant compte des préoccupations exprimées par nos deux assemblées. Avec le président Buffet et Marc-Philippe Daubresse, nous avons tenu un certain nombre de points durs dans cette négociation.

est une bonne nouvelle pour le Parlement, en particulier pour le Sénat. La Haute Assemblée a pu apporter à ce texte des ajouts robustes juridiquement, tirés de l'expérience et des remontées de terrain des collectivités territoriales, que nous représentons, avec une vraie exigence de préservation des libertés publiques.

d'abord dans nos maires et nos polices municipales : nous voulons faire confiance aux élus de terrain ; nous voulons donner la possibilité, avec l'article 1, à ceux qui le souhaitent de faire expérimenter des compétences nouvelles à leurs agents, dans le strict respect de leurs compétences et de celles de l'État. Nous avons pu entendre ici ou là dans les débats que cet article marquerait une forme de désengagement de l'État ou qu'il aboutirait à confier des missions régaliennes à des agents de police municipale n'étant pas en capacité de les exercer. Je tiens à le redire ici solennellement, l'ambition du Gouvernement, qui rejoint celle des rapporteurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, est bien une ambition de multiplication territoriale de la sécurité et en aucun cas de régression. L'enjeu pour nous est bien de donner des moyens nouveaux aux forces municipales et de permettre à ceux qui le veulent de pouvoir mieux répondre aux troubles du quotidien. J'ai été élue locale, comme vous, et je sais combien il peut être frustrant de ne pas pouvoir agir sur les nuisances de tous les jours qui empoisonnent la vie de nos administrés. Ce texte nous permet de dire aux élus qui le souhaitent : « Allez-y Partir du principe que nos agents de police municipale ne sauraient pas faire témoigne, à mon sens, d'une conception curieuse de cette troisième force à l'heure où elle s'affirme plus que jamais comme un partenaire essentiel des forces de sécurité intérieure. J'en profite pour rendre hommage

et valorisant les polices municipales, le texte renforce l'intérêt pour les communes de s'en doter. Il n'est nul besoin ici de rappeler l'article 4, qui ne permet rien moins que de créer à Paris la plus importante police municipale de France. Pour pallier les difficultés des communes à se doter d'une police municipale, l'article 5 renforce les possibilités de mutualisation à l'échelon intercommunal comme cela n'avait jamais été fait auparavant : SIVU, Sivom, EPCI à fiscalité propre, contrat de mise à disposition. Par ailleurs, l'article 20 A va permettre la mutualisation des dispositifs de vidéoprotection dans le cadre d'un centre de supervision urbain réunissant l'ensemble des parties prenantes. Bref, tout est fait pour doter les maires de capacités à véritablement mettre en oeuvre une sécurité du quotidien.

sur les drones et les caméras embarquées, auxquels les policiers municipaux vont désormais pouvoir avoir recours pour les compétences que le législateur leur attribue, dans cette seule limite- nous en avons débattu en évoquant les libertés récemment -, et évidemment à chaque fois en coordination avec les forces de sécurité intérieure. Confiance Confiance ensuite dans notre secteur privé de sécurité : la grande réforme de refonte sans précédent du cadre de la sécurité privée que nous menons ne trahit aucune défiance de notre part. Au contraire, elle vise à accompagner ce secteur, qui est en pleine expansion, et à lui donner et à lui donner les moyens d'être pleinement reconnu comme un partenaire de confiance. Cette confiance a évidemment pour contrepartie la responsabilisation des acteurs de ce domaine. Charge à eux désormais d'assurer cette montée en compétences et en moyens, notamment en vue des grands rendez-vous qui sont devant nous, comme la Coupe la Coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques de 2024. Confiance aussi dans la force du lien qui unit la police et les citoyens : cette confiance s'exprime dans la mise en place, grâce à l'article 27 - c'est une mesure que nous appelons de nos voeux dans le cadre du Beauvau de la sécurité -, d'une réserve opérationnelle de la police nationale alignée sur celle, ô combien efficace, de la gendarmerie nationale. Elle pourra répondre, avec des missions rénovées, à la demande très forte d'engagement des Français et à la volonté que nous avons avec le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, de valoriser la police nationale et de continuer à la faire bénéficier de la compétence de réservistes toujours plus nombreux, aux profils plus variés et aux engagements plus divers. Elle permettra de maintenir dans les cinq années après leur départ la qualification d'officier de police judiciaire pour les retraités ayant bénéficié de cette qualité pendant leur carrière. Cette évolution, soutenue par le sénateur Henri Leroy, que je salue, constitue une avancée forte et appréciée. Il s'agit également d'un texte de protection de nos forces. Les moyens vidéo, notamment les drones- j'y insiste -, démultiplient les capacités d'action des forces en les exposant moins aux dangers de voie publique ou en leur permettant de porter secours dans des conditions d'exercice parfois terriblement complexes et dangereuses. Le Sénat a encadré leur usage de nombreuses garanties, dont il nous appartiendra désormais d'assurer la déclinaison la plus opérationnelle possible et, bien entendu, la plus respectueuse des libertés. Je constate par ailleurs avec satisfaction que les parlementaires des deux chambres partagent pleinement la volonté du Gouvernement de protéger spécifiquement les policiers et les gendarmes. Ainsi, les articles 23, sur les crédits de réduction de peine, 23 , sur l'extension du délit d'embuscade, 24, qui prévoit un délit de provocation à l'identification, mais également 27 , qui étend la protection fonctionnelle à l'audition libre pour les membres des forces de sécurité intérieure, sont autant de dispositions qui viennent témoigner de l'attention particulière de la République envers ceux qui la protègent. s'agit enfin d'un texte de fermeté. Fermeté vis-à-vis de ceux qui brisent des vies par leur comportement irresponsable sur la route, en assouplissant les possibilités de contrôle de l'alcoolémie ou de la consommation de stupéfiants. Fermeté vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas les règles dans les transports : nous avons introduit une disposition qui permettra de renforcer substantiellement les moyens d'action des opérateurs du secteur pour lutter contre la fraude, tandis que les possibilités en matière de recours vidéo sont par ailleurs renforcées dans la loi. Fermeté aussi pour mieux encadrer les produits dangereux, comme les mortiers : cela a été débattu. Fermeté, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot. Je sais que vous êtes toutes et tous ici favorables à ce que l'État de droit républicain soit respecté. Au final, avec le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, nous souhaitons véritablement saluer la hauteur de vues des débats et la très grande qualité du travail de MM. les rapporteurs lors des auditions, de l'examen en commission des lois, puis en séance. Certes, le Gouvernement regrette que les règles strictes de l'article 45

de compromis. C'est avec le même esprit de consensus et de sagesse républicaine que je vous invite à examiner et à voter le texte qui vous est soumis et auquel le Gouvernement n'apportera, comme c'est l'usage, que de simples amendements de coordination et d'application en outre-mer. La parole

On peut souscrire à l'idée d'une coordination des forces de sécurité nationales, municipales et privées en vue de grands événements, comme la Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques. Mais, pour nous, ce texte semble à contretemps, enchâssé entre le Livre blanc de la sécurité intérieure, le Beauvau de la sécurité et la future loi d'orientation. Débattre d'un nouveau cadre légal d'usage des drones et des caméras embarquées ou de captation des images par les forces de sécurité aurait à nos yeux mérité une expertise plus approfondie et un débat public préalable. Au final, la proposition de loi, qui visait initialement à la mise en adéquation des polices municipales et de la sécurité privée à partir du concept de continuumde sécurité, se traduit par un texte avec des mesures disparates qui affectent la lisibilité et la sécurité juridique des principales dispositions. Je souhaite évoquer quatre difficultés. Premièrement, concernant les polices municipales, nous nous opposons au champ trop étendu de l'expérimentation, qui pourrait, contrairement à ce que vous indiquiez, madame la ministre,

notamment sur la sous-traitance, au risque d'aboutir à des prestations à la baisse et de précariser le personnel. Outre les habilitations données au Gouvernement visant l'organisation du Cnaps et la formation pour l'accès à la profession, plusieurs dispositions posent des difficultés de nature constitutionnelle. Je pense au rétablissement à cinq ans de la durée nécessaire de détention d'un titre de séjour pour qu'un ressortissant étranger puisse exercer dans le secteur, au fait de confier des missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes aux agents de sécurité privée ou encore à la suppression de l'habilitation spécifique de l'agrément pour réaliser des palpations de sécurité. Troisièmement, les dispositions relatives à la vidéoprotection

Nous restons opposés à la quasi-totalité des mesures inscrites dans le titre III. Elles sont manifestement contraires à la Constitution, en particulier au principe de protection de la vie privée. Nous récusons l'évolution de la doctrine d'emploi des caméras-piétons, qui vont devenir des accessoires du maintien de l'ordre public alors qu'elles avaient plutôt pour objet initial de sécuriser les agents ou d'apaiser les relations entre la police et la population. Nous ne comprenons pas le rétablissement par la commission mixte paritaire des mesures élargissant les possibilités de déport d'images et de vidéosurveillance, notamment dans les halls d'immeuble. De même, la possibilité pour la RATP et la SNCF d'avoir accès aux images de vidéoprotection dénote quelque part un glissement d'une mission de surveillance à une mission régalienne. De manière globale, les dispositifs relatifs à la création et et l'encadrement des régimes légaux intéressant l'usage des drones et des caméras embarquées soulèvent des interrogations pour nous. Quatrièmement, les dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure nous interpellent. s'est accordée sur une réécriture technique de l'article 24 qui laisse entière la menace contre la liberté de la presse et renforce les sanctions

Même difficulté avec l'article 23, qui supprime les crédits de réduction de peine et l'automaticité des remises de peine. Enfin, nous restons opposés à l'autorisation de port d'arme pour les policiers et gendarmes hors service dans les établissements recevant du public.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la chronologie de la navette parlementaire est bouleversée par le télescopage des articles 24 de cette proposition de loi pour une sécurité globale et 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, que nous sommes en train d'examiner depuis quelques jours. Ces deux articles ont sensiblement le même objet, à savoir protéger les forces de l'ordre des captations malveillantes d'images, mais ils sont présentés simultanément dans deux véhicules législatifs. On se On se souvient aussi de la volonté du Gouvernement de créer une commission à sa mesure pour une nouvelle écriture de l'article 24 ... Ce grand n'importe quoi, alors que les Français attendent de la clarté, met en lumière le mépris de l'exécutif pour la démocratie représentative. Un texte de sécurité globale doit garantir une sécurité démocratique avant tout, sans quoi on bascule dans un régime aux pouvoirs démesurés. Le rôle de l'État est de garantir aux citoyens et aux collectivités la liberté et la sécurité ! La réalité montre que l'insécurité se généralise, tout autant que le recul de nos libertés. Perdue, La République En Marche se met à courir et se prend les pieds dans les marches. Nous avons ici la preuve, au mieux, de la mauvaise communication, au pire, du désaccord entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice. Chacun porte sa mesure dans son coin, et les Français, qui attendent une conjonction des réponses policières et pénales, en sont les premières victimes. S'agit-il d'une lutte d'ego, d'un combat de coqs, d'une divergence nette de ligne ou d'une stratégie qui mettrait en scène le duo du méchant et du gentil pour satisfaire tout le monde ? Que l'on examine la loi dans de telles conditions est déjà insupportable ; mais passe encore ... Le pire est que ce cafouillage affiché met à mal la crédibilité de l'État, alors que celui-ci a tant besoin de retrouver sa légitimité et son autorité. Et dire que, du locataire de Beauvau à celui de la Chancellerie, ce sont les mêmes qui ne manquent jamais une occasion de faire la leçon sur le prétendu manque de sérieux et de cohérence des parlementaires, avec un dédain affiché pour les communes À ce stade, je préférerais pourtant donner la boussole et les manettes à nos communes plutôt qu'au Gouvernement, car elles aussi attendent que l'on apporte des solutions ciblées aux problèmes de sécurités locales. Ce grand n'importe quoi devrait entraîner le rejet des conclusions de la commission mixte paritaire en attendant que le Gouvernement accorde ses violons. Les sénateurs, représentant des élus de la réalité des terroirs et des territoires, étaient en droit d'obtenir un peu plus de respect.

L'adoption d'un nouveau texte visant à assurer une sécurité globale tout en préservant les libertés était malheureusement nécessaire, car nous assistons depuis de nombreuses années à une nette dégradation du climat sécuritaire dans notre pays. Les actes de violence se multiplient, notamment contre nos policiers, nos gendarmes et nos pompiers. Il est donc indispensable de mieux protéger les fonctionnaires qui participent à une opération de police contre tous ceux qui se permettent de dévoiler leur identité. Grâce à la sagesse du Sénat, la nouvelle rédaction de l'article 24 y parvient. Si cet article avait fait l'objet de nombreuses controverses, sa nouvelle rédaction clôt les polémiques en remplissant l'objectif de protection sans pour autant porter atteinte à la liberté de la presse. Je tiens aussi à le rappeler, les forces de l'ordre ne sont pas les seules concernées. Les élus sont eux aussi trop souvent visés par des violences inadmissibles. La vocation de nos forces de l'ordre est de protéger les Français, celle des pompiers ou des médecins de leur porter secours et celle des élus de Quel triste retournement du devoir : protéger ceux qui nous protègent ! Car, au-delà des victimes directes, ces attaques portent aussi atteinte à l'ensemble de la République et à la cohésion de notre société. Il est grand temps que cela cesse. Ces dispositions s'accordent d'ailleurs avec la promesse qu'avait formulée le Premier ministre lorsqu'il avait assuré solennellement devant le Sénat et le pays qu'il n'y avait pas et qu'il n'y aurait pas de zone de non-droit sans contrôle d'identité. Nos concitoyens attendent légitimement un renforcement de la sécurité. Les dispositions figurant dans ce texte permettront de donner davantage de moyens aux forces de l'ordre dans l'accomplissement de leur mission. mission. Ainsi, la vidéoprotection sera étendue, afin de permettre à cette technologie de déployer tous ses effets. Comme toujours, le Sénat a prêté une attention particulière à la protection des libertés publiques.

après avis de la CNIL. Cette nouvelle garantie renforcera encore la protection des libertés de nos concitoyens. À côté du secteur public, le secteur privé constitue un important pilier du continuum de sécurité. La proposition de loi que nous examinons renforce le contrôle de la sous-traitance. Elle contribuera à améliorer la qualité des prestations et la légitimité des sociétés qui les exécutent. Ce texte prévoit également une expérimentation visant à confier des prérogatives de police judiciaire à certaines polices municipales.

à quinze agents. Je voudrais redire ici avec force à quel point il est essentiel de s'assurer que les petites communes ne sont pas pénalisées. Le législateur doit veiller à ce que la sécurité soit uniforme sur l'ensemble du territoire. Cela implique de tenir compte du fait que les petites communes n'ont pas les moyens de recruter des agents de police municipale. En définitive, c'est donc à l'État qu'il revient en premier lieu d'assurer la sécurité de nos concitoyens. dispositions de ce texte concourent à améliorer la sécurité des Français. Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de son adoption, tout en rappelant que la question des moyens financiers consacrés à nos forces de l'ordre reste fondamentale pour parvenir à nos fins.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, entre états d'urgence sanitaire et sécurité globale, la succession de textes

loi prône la surveillance de masse, de la légalisation et de l'extension de l'usage des drones au plus grand déploiement des caméras-piétons, sans préciser, pour ce dernier outil, l'importance du contrôle de l'action de l'agent dans le cadre de ses fonctions. Il aurait évidemment été judicieux d'inscrire dans la loi que cette technologie a pour objet principal le renforcement de l'action de la justice et l'aboutissement des plaintes des victimes de violences commises par certains agents. Ce texte s'attaque à la liberté d'expression, en limitant la dénonciation des actes répréhensibles des forces de l'ordre, par son article 24. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme le souligne : l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression doit répondre à un besoin social impérieux. Or, comme le relève l'avis de la Défenseure des droits, l'infraction initialement prévue n'était pas nécessaire à la protection des policiers et gendarmes. Malgré sa réécriture, la critique faite à cet article ne semble pas pour autant obsolète. La proposition de loi porte également une atteinte disproportionnée à la liberté d'informer. Le nouveau délit de provocation à l'identification, une notion floue, ouvre la voie à des interprétations divergentes et arbitraires pouvant nuire au travail des journalistes. Ce sont ces images, diffusées dans la presse, qui ont permis de rendre publique, par exemple, l'affaire Benalla, n'en déplaise au Gouvernement. Ce texte bride le droit de manifester, parce qu'il crée un climat anxiogène autour des manifestations publiques. Il légalise les drones, mais reste silencieux quant aux LBD et grenades de désencerclement, que nous savons pourtant être la cause de nombreuses blessures et mutilations. Alors, « préservant les libertés », dites-vous ? Voilà une appellation assez antinomique, si je puis me permettre Enfin, nous sommes pour la création d'une police municipale à Paris. Nous nous associons à la vision que la mairie de Paris a de sa future police municipale une police de proximité formée aux questions sociétales et à l'image de ceux qu'elle protège. Alors, votez ce texte ! Mais nous sommes contre le dangereux rapprochement qu'opère ce texte des prérogatives et statuts de la police et de la gendarmerie nationales, de la police municipale et de la sécurité privée. Force est de constater que ce texte ne s'appuie sur aucune vision réellement novatrice et complète de la sécurité en France. Il n'a, hélas ! de global que le nom. Pour ces raisons, le groupe Écologiste- Solidarité et Territoires votera contre. C'est dommage

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, compte tenu de l'inspiration de cette proposition de loi et de l'attitude des forces politiques au sein de notre assemblée comme de l'Assemblée nationale,

professionnels partagés entre police, gendarmerie et police municipale, de nombreux progrès ont été accomplis. Au fond, la reconnaissance de la capacité des polices municipales à devenir les contributeurs d'une sécurité plus active,

Je peux vous dire que l'on partait de loin ! La prévention, dans la société française, contre ces sociétés et la très grande méfiance qui les entourait ont demandé un certain effort à la majorité de l'époque- je peux en témoigner

permettant de mettre en place un système de vidéosurveillance dans l'espace public, avec un contrôle organisé,

est vrai que nous aurions souhaité aller plus loin dans la régulation des sociétés privées en matière de contrôle de la sous-traitance ou de la qualité des formations proposées. Sur les caméras aéroportées, le texte prévoit également, grâce à l'apport du Sénat, de fixer des cadres d'usages, comme de réaffirmer la prohibition de techniques telles que la captation des sons, la reconnaissance faciale, les interconnexions automatisées de données. Il nous appartiendra de suivre très régulièrement la pertinence de ces dispositions et de les réadapter en conséquence au regard des pratiques qui évoluent plus vite que le droit. Je compte ici prendre rendez-vous avec mes collègues du Sénat au moment de la discussion du budget, pour qu'ils permettent à la CNIL d'assurer pleinement la montée en régime et la diversification de ses missions. Il appartient en effet à la puissance publique de pouvoir organiser les contrôles adéquats. adéquats. Je réaffirme ici notre attachement viscéral à ce que le cadre de travail de nos forces de l'ordre et forces de sécurité prenne appui sur nos libertés fondamentales : usage proportionné et délimité strictement aux missions et aux temps de ces missions, respect des libertés individuelles et de la presse. C'est notre fil rouge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une majorité du groupe du RDSE continue de s'opposer à la détention possible d'armes par des forces de l'ordre hors service au sein d'établissements recevant du public. J'en viens à une interrogation majeure relative aux dispositions liées aux expérimentations de mise en commun entre les communes de policiers municipaux. Quelques dispositions de notre groupe ont été adoptées comme la nécessité d'un débat au sein de chaque commune expérimentant les polices intercommunales, la publication des frais de formation engendrés par cette réforme ou l'élargissement des pouvoirs de verbalisation des gardes aux espaces naturels non boisés. Dans l'ensemble, ces expérimentations appellent quelques réflexions. Non, la police intercommunale nouvellement créée ne saurait être une troisième force de sécurité ! Nul ne comprendrait que cette réforme soit un prétexte au désengagement de l'État.

L'aménagement du territoire que nous défendons exige une intervention publique constante qui vient corriger des déséquilibres, inscrit la force publique dans tous les territoires, y compris ruraux, de France périphérique et d'outre-mer. l'expérimentation est un outil formidable, elle touche en l'occurrence à la sécurité des biens et des personnes et elle durera cinq ans. Ce n'est pas rien ! Après cinq ans, il sera très difficile de revenir en arrière. Aussi, nous demandons une évaluation rigoureuse, y compris à l'échelon local.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « La France- berceau des droits humains tels que promulgués en 1789 -serait-elle en train de rejoindre le camp des pays où la démocratie est fragilisée par le pouvoir lui-même ?

Avec eux, nous nous inquiétons du « recul de la démocratie » dans le monde et en France, en pleine pandémie, à l'heure où les populations souffrent d'un recul global des droits humains et des libertés. Je vous le dis solennellement : aujourd'hui, en posant un point final aux débats parlementaires autour de ce texte, nous actons un recul sans précédent de nos libertés publiques. L'État affirme son autorité et la remise en cause de celle-ci ne sera que très peu tolérée Des mobilisations importantes ont permis une réécriture du si problématique article 24. Mais quelle réécriture ? Ne soyons pas dupes. Si la question de l'« usage malveillant de l'image », qui posait de sérieuses difficultés dans la démonstration de l'intentionnalité, a été résolue, la formulation finale de l'article visant une « provocation à l'identification » qui a pour objectif « manifeste » de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers ou des gendarmes ne pose pas moins question. Comment prouver ou non ce but manifeste quand une image est diffusée pour dénoncer un comportement de violence policière, par exemple bien d'autres mesures qui seront aujourd'hui définitivement adoptées mériteraient que ce texte soit purement et simplement retiré. En commission mixte paritaire, les arbitrages se sont révélés anecdotiques, puisque la philosophie globale de ce texte était partagée d'emblée par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale et par la majorité de droite au Sénat. leur objectif d'instaurer un « continuum de sécurité » allant des policiers nationaux aux policiers municipaux, en passant par les gardes champêtres et les agents de sécurité privée. Quelques contraintes sont instaurées pour encadrer les entreprises de sécurité privée, en échange de quoi les agents de sécurité privée se voient accorder de nouveaux pouvoirs ils pourront être autorisés par le préfet à effectuer des missions de surveillance de la voie publique dans le cadre de la lutte antiterroriste. Qui plus est, ils n'auront plus besoin d'habilitation pour procéder à des palpations de sécurité dans le cadre de certaines manifestations. Comment octroyer de tels pouvoirs à des entreprises qui, par définition, n'ont qu'un but marchand ? De nouveaux pouvoirs sont également transférés aux polices locales, sous la tutelle des maires, lesquelles se substituent de plus en plus à la police nationale sans en avoir ni les moyens ni les formations requises. Nous l'avons signalé à plusieurs reprises lors de l'examen du texte : à ce maillage fin du territoire en matière d'agents de sécurité se couple une extension démesurée de l'usage des nouvelles technologies. Certes, la commission des lois du Sénat s'est efforcée d'encadrer les dispositifs proposés, notamment en matière d'usage des drones, mais cela est largement insuffisant. Nous entrons désormais dans une nouvelle ère en matière de surveillance des populations, ce que nous ne pouvions soupçonner voilà encore quelques années. Aujourd'hui, il s'agit uniquement de « capter des images », nous explique-t-on. Qu'en sera-t-il demain ? Si les garanties sont aussi faibles et éphémères que celles qui ont été apportées à la loi SILT de 2017, alors le pire est à craindre, et cela n'a rien d'alarmiste que de le dire. Gageons que les Sages du Conseil constitutionnel, qui seront saisis, vous feront, eux, entendre raison. Pour l'heure, mes chers collègues, prenons la mesure de ce qu'implique notre vote aujourd'hui pour notre pays, pour la sauvegarde de nos libertés et droits fondamentaux, et opposons-nous à ces conclusions.

la proposition de loi sur laquelle nous sommes conduits à nous prononcer a suscité, rappelons-le, d'importants remous dans le débat public et donné lieu à de nombreuses manifestations sur la voie publique en dépit même des contraintes particulières tenant à la crise sanitaire. Aussi, c'est avec un certain soulagement que nous nous apprêtons à voter en faveur du texte de compromis sur lequel se sont accordés députés et sénateurs, le 29 mars dernier. Que de chemin parcouru avant d'aboutir à cet accord ! Rappelons-nous : dès le mois de décembre 2020, peu après l'adoption du texte en première lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat, pris en la personne de nos deux chers rapporteurs, a fait part de sa vive détermination à améliorer l'article litigieux, le « fameux » article 24. Notre groupe s'est en outre vigoureusement opposé à la désignation d'une commission nommée spécialement pour réécrire cet article, rappelant

Cette opposition fut féconde, puisque la version sénatoriale de l'article 24, élaborée sur l'initiative de la commission des lois, a fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées en commission mixte paritaire. D'importantes garanties y ont été apportées. L'ultime version a totalement abandonné toute référence à loi de 1881 sur la liberté de la presse, tout en maintenant l'objectif initial par la création d'un nouveau délit de provocation à l'identification des policiers, et ce dans un but manifeste de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Ce délit sera dorénavant inscrit dans le code pénal. Il s'agit d'une réécriture plus sûre d'un point de vue juridique. Cette nouvelle rédaction ne porte pas atteinte à la liberté de la presse et lève toute ambiguïté sur une prétendue pénalisation d'intention. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Outre le volet de cet article très controversé, de nombreuses modifications sénatoriales ont été conservées dans le texte que nous examinons. Sans revenir

éligible aux seules communes qui emploient au moins vingt agents de police municipale, le Sénat a ouvert cette possibilité aux communes qui disposent d'au moins quinze agents. De plus, dans un souci de cohérence, le Sénat a souhaité que cette expérimentation soit prévue non pas pour une durée de trois ans, mais pour une durée de cinq ans, afin d'en calquer la durée sur celle du mandat municipal en cours pour en mesurer pleinement tant l'intérêt que les effets. Notre volonté de mieux protéger ceux qui nous protègent nous a conduits à renforcer les peines encourues en cas de violences commises en raison de leurs fonctions sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Ces peines seront également applicables en cas de violences commises sur leurs proches. Par ailleurs, face à la multiplication des intrusions dans les exploitations agricoles, régulièrement visitées, cambriolées ou dégradées, le Sénat a élargi les prérogatives des policiers municipaux et des gardes champêtres en les autorisant à constater le délit d'intrusion illégale dans une exploitation De nombreuses garanties ont également été apportées par le Sénat aux technologies de vidéosurveillance et de captations d'images, garanties particulièrement nécessaires au regard des risques qu'elles présentent en termes de libertés individuelles comme de libertés publiques. Si nous devions émettre un regret, c'est la disparition des dispositions adoptées par le Sénat, sur proposition de Dominique Estrosi Sassone, qui entendaient clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation. Elles auraient sans doute permis de renforcer la jouissance paisible des propriétaires et locataires. Malgré cela, nous nous réjouissons que les dispositifs souhaités et votés par la majorité sénatoriale en faveur de la sécurité, pour lesquels nous avons pris soin qu'ils ne s'accompagnent pas d'un désengagement de l'État, aient largement retenu l'attention de la majorité à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, je tiens à remercier chaleureusement le président de la commission des lois, cher François-Noël Buffet, et nos deux excellents rapporteurs, Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, qui, malgré les zones de turbulences rencontrées par ce texte, n'ont commis aucune erreur de navigation. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur le bien-fondé et l'utilité du bicamérisme, l'enrichissement par le Sénat de ce texte apporte une réponse sans ambiguïté. Pour l'ensemble de ces raisons exposées, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi élaborée par la commission mixte paritaire. La parole

avec conviction. Le Sénat s'était assigné comme objectif de dépasser frénésie et posture pour adapter la loi aux évolutions de la délinquance et de la violence, mais aussi aux évolutions des nouvelles technologies, lesquelles peuvent aussi aboutir par l'image à menacer ceux qui nous protègent, les transformant en cibles et parfois, trop souvent déjà, en victimes tragiques. Chacun de nous pense ici aux représentants des forces de police et de gendarmerie qui, parce qu'ils nous protégeaient,

par une loi ciselée et sécurisée juridiquement, voire apaisée sur l'article 24, qui a soulevé tant d'opprobre. L'article 24 est donc désormais cicatrisé. Il ne touche plus à la loi de 1881 sur la liberté de la presse et crée un nouveau délit de « provocation à l'identification » des policiers, qui saura trouver sa place dans la protection de nos forces de l'ordre. Au cours de nos débats, j'ai appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur

à celle de la police nationale ou de la gendarmerie, car, il faut le rappeler, l'État doit assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire ; les polices municipales gèrent la tranquillité du voisinage. En cela, je salue les initiatives très positives des rapporteurs sur la mutualisation des polices municipales.

et s'inscrit dans l'avenir. Reste une alerte que je me dois de vous adresser, madame la ministre, sur l'expérimentation de l'article 1 visant l'extension des prérogatives des polices municipales. Le principe de cette expérimentation est une excellente chose, répond à un besoin

visant à garantir le principe de libre administration des communes et à empêcher que ne soit imposé de manière verticale et autoritaire un futur transfert

que chat échaudé craint l'eau froide. Cette expérimentation doit sécuriser, après son évaluation exigeante, un principe d'élargissement de ses compétences aux seules collectivités volontaires.

l'un des piliers de notre démocratie. J'espère que nous aurons su, par ce texte, apporter des solutions aux peurs qui se font jour dans la population et renforcer la protection de ceux qui nous protègent. La discussion

modeste, afin d'introduire la notion de pluridisciplinarité dans l'enseignement des faits religieux. L'expression « fait religieux » a été proposée par Régis Debray dans un rapport rendu au ministre de l'éducation nationale en 2002. en 2002. Il y insistait bien sur le fait que « l'histoire des religions [ ...] ne saurait prétendre, au lycée et au collège, occuper une place à part. La charge en incombe aux personnels en fonction, à travers les disciplines reconnues ». Je crois qu'il est extrêmement important de dire

de la culture ? Les discussions autour d'un enseignement des faits religieux sont fortes au sein de l'éducation nationale depuis la remise du rapport Debray sur le sujet en 2002.

qu'en histoire les élèves sont amenés à étudier, dans l'ordre chronologique, les religions juive, chrétienne et musulmane.

avons besoin d'avancer sur cette question. Or le sens de votre amendement, c'est justement de renforcer ce que nous avons souhaité mettre en place, en insistant sur la dimension pluridisciplinaire.

C'est pourquoi j'ai fait cette remarque sur l'histoire. Ce n'est pas simplement un débat de spécialistes ou un débat théorique : c'est une question vraiment importante. Pour ma part, je considère que la pensée d'Edgar Morin sur ce sujet est très juste, mais qu'elle ne doit pas être mal interprétée : elle consiste à insister sur la complexité

qui me semble résumer la totalité de ce que nous voulons mettre en avant : « Il serait sage [ ...] de considérer que les " faits religieux " ne sont pas enseignés pour eux-mêmes, mais présentés et explicités dans le cadre d'enseignements pluridisciplinaires qui les mobilisent.

parents-école est au coeur des problématiques sur les inégalités et la réussite scolaire en général. Les enfants les plus en difficulté sont souvent ceux qui ont les parents les plus éloignés du système éducatif, car ils sont parfois pénalisés par la faible compréhension des attendus scolaires, de l'éducation civique, de la citoyenneté.

parents. Dans ce type d'échanges, les parents peuvent intégrer des idées qu'ils ignoraient parfois, comme la laïcité et les valeurs républicaines portées par l'école publique. Il est nécessaire de créer une « alliance éducative » entre parents et enseignants, dans l'intérêt de l'enfant et de la République. Tel est le sens de cet amendement.

les enseignants et les parents, qui ont fortement évolué depuis quelques années. Les enseignants ont sans doute besoin d'outils de formation

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Yves Roux. Le présent projet de loi fait de la laïcité l'un des leviers fondamentaux de lutte contre les séparatismes, notamment en milieu scolaire. Dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, présidée par notre collègue

Dans cet esprit, l'amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l'espace scolaire en la faisant signer par les enseignants et les parents d'élèves. Il s'agit de réaffirmer que la laïcité, comme les principes républicains, contribue à la formation de citoyens éclairés, dans le respect de la diversité des croyances

Dans cet esprit, le présent amendement vise à promouvoir la charte de la laïcité dans l'espace scolaire, en exigeant son affichage de façon visible dans tous les établissements du premier et du second degrés, qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Lors de l'examen de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, nous avons gravé dans notre droit la présence obligatoire du drapeau français, du drapeau européen et des paroles de l'hymne national dans toutes les salles de classe. Notre proposition s'inscrit dans le droit fil de cette initiative de valorisation de nos symboles de rassemblement. Nous souhaitons également que la laïcité, qui est au coeur du pacte républicain, figure en bonne place dans nos écoles. La laïcité est au fondement de notre système éducatif depuis la fin du XIX siècle ; elle permet de protéger les élèves du prosélytisme et des emprises idéologiques. Cela passe par un apprentissage permanent des règles du vivre ensemble que prône la charte de la laïcité. L'éducation nationale, dans son organisation publique ou privée, s'attachera ainsi à former des citoyens éclairés qui s'épanouiront dans le cadre commun de principes républicains.

provient très largement de l'enseignement de la laïcité auprès de notre jeunesse. Dans toutes les écoles, publiques et privées, la laïcité ne peut ni ne doit être mise de côté,

Cela signifie que le chef d'établissement, sur la seule base de sa suspicion, pourra remettre en cause un certificat médical, pourtant établi par un médecin.

Certes, il faut peut-être se saisir de la question des certificats de complaisance, mais il s'agit ici d'une question relative à la perception de la pratique du sport, ainsi qu'au rapport au corps et à l'exercice physique en collectivité. Il s'agit moins souvent d'une question de respect des principes républicains que d'une question de santé publique et de rapport au sport. Nous sommes favorables à ce que cette question soit traitée, mais de manière apaisée, de la proposition de loi relative au sport, qui devrait avoir lieu dans quelques mois. Développer la pratique sportive grâce à l'école est un objectif important de santé publique. Si vous étiez réellement attachés à la question de l'évaluation médicale de la pratique sportive, vous feriez mieux de commencer par allouer des moyens au recrutement d'un nombre accru de médecins scolaires, qui font tant défaut aujourd'hui. Cet article ne saurait se résumer à une mesure d'affichage.

déjà ceci : « L'EPS fait partie des disciplines pour lesquelles les professeurs se plaignent souvent de manifestations ou d'interventions de nature religieuse perturbant leur enseignement. » Ce constat a été conforté par la mission de l'inspection générale

Le sport véhicule les valeurs de fraternité et d'égalité indispensables au vivre ensemble, tandis que la culture est l'un des vecteurs d'une bonne intégration sociale. Nos écoles, soutenues par les collectivités locales, s'emploient à faire accéder les enfants au sport et à la culture en marge du programme obligatoire. Afin de rassembler tous les enfants et pour contribuer à les brasser de manière à favoriser la mixité sociale, nous proposons, par cet amendement, d'encourager les inspecteurs d'académie à veiller à ce que soient associés les enfants d'une même classe d'âge des établissements privés hors contrat ou sous contrat avec l'État aux activités sportives et culturelles périscolaires.

les comportements portant atteinte à la mixité entre filles et garçons en font partie. Dans certaines écoles, des enseignants ont pu observer des filles et des garçons se tenir volontairement à distance dès leur plus jeune âge. Comme le rappelle souvent le Gouvernement dans le cadre de sa politique éducative, l'égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le code de l'éducation. Son respect encourage un cadre scolaire serein et protecteur et l'apprentissage de l'interdiction des violences sexistes. Au-delà, il s'agit de favoriser l'égalité en matière d'orientation. Aussi, cet amendement vise à ce que ce principe soit respecté dès l'école, en impliquant pour ce faire le conseil d'école. le conseil d'école. Celui-ci rassemble la communauté éducative de l'établissement, les collectivités locales et les représentants des parents d'élèves ; il doit être un outil de transmission des informations sur les éventuels manquements à l'égalité entre les hommes et les femmes.

de l'éducation nationale. Le présent amendement vise à étendre la destination des certificats médicaux au directeur d'école ou au chef d'établissement. En effet, on sait que le certificat médical est donné directement au professeur d'éducation physique et sportive, voire au CPE.

La cantine est un passage important dans la vie d'un écolier : il y prend ses premières marques par rapport aux règles de tenue en société et y découvre les prémices de la tradition culinaire française. ce modèle est en péril, car l'alimentation est devenue l'une des cibles privilégiées des séparatistes et des islamistes. En outre, de plus en plus d'écoles font face à des demandes religieuses, telles que des menus sans porc, ou sont sommées d'abandonner toute viande qui ne soit pas halal. Les revendications de ce type posent plusieurs problèmes. Avant tout, elles créent des divisions chez les enfants, au risque de mettre à part ceux qui mangeraient du porc, quand ils deviennent minoritaires. Peu à peu, l'exception devient la généralité, au point que, dans de nombreux quartiers, le terme de « séparatisme » ne convient pas pour définir la réalité : il s'agit plutôt d'un remplacement qui se développe dès le plus jeune âge. revendications posent aussi un problème de coût, d'organisation et de principe pour les communes. Les maires sont souvent désemparés face à ce problème : la loi ne les soutient pas assez. Ils sont alors exposés à des pressions, voire à des accusations. D'autres élus, au contraire, en profitent pour agir par idéologie ou électoralisme, parfois même sous couvert d'écologie. La décision récente de la mairie de Lyon de mettre en place des repas sans viande toute l'année illustre parfaitement ce renoncement progressif à proposer du porc ou toute viande qui ne soit pas homologuée par les islamistes. est contraire à tout intérêt culinaire, nutritionnel, ou écologique : c'est l'idéologie communautariste soutenue par les talibans verdoyants et servie dès le plus jeune âge dans les assiettes Les revendications communautaires se multiplient : pétitions, plaintes des parents et pressions diverses. Face à cela, la loi doit soutenir les maires et rappeler qu'elle défend l'égalité à l'école et non la distinction. Les cas de renoncement sont multiples, ils ne sont pas seulement l'apanage de la gauche en 2012, Édouard Philippe, alors élu au Havre, avait fait jeter 8 500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires, parce qu'elles contenaient de la gélatine de porc ! Les menus sans porc ou sans nourriture halal, ainsi que toute autre pratique visant à appliquer à l'école publique française des principes religieux, doivent être prohibés dans notre pays. Avez-vous déjà entendu des polémiques demandant du poisson le vendredi ? Certainement pas ! Ce sont toujours les mêmes qui sont derrière les provocations : les islamistes ! Il faut les nommer, faute de quoi on ne pourra pas avancer. Cet amendement a donc pour objet de répondre à une vraie demande des parents d'élèves, des directeurs d'école et des maires, au nom de l'intérêt supérieur de l'élève, afin d'éradiquer les germes de l'islamisme dans l'école publique.

dans les dérives que vous évoquez. Par ailleurs, je m'interroge sur la qualification de « repas confessionnel » : qui va déterminer s'il s'agit ou non d'un repas confessionnel ? Pour ces différentes raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel

On n'interdit pas un fantasme ; ce n'est pas par un amendement qu'on guérit une obsession ! Si on entend par « menu confessionnel » des menus halal ou casher, il faut savoir qu'ils n'ont jamais été imposés dans les écoles publiques françaises, alors que le sujet est régulièrement agité dans le débat politique. En 2012, il dix ans, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen annonçait vouloir interdire le halal dans les cantines françaises, faisant accroire que de tels menus étaient servis ; c'était déjà faux. Dix ans de mensonges, donc ! Régulièrement, à toutes les élections, le débat revient sur la table, si je puis dire. Ce que proposent de nombreuses cantines, ce ne sont pas des menus confessionnels, mais un choix : la possibilité d'un repas sans viande, dit « de substitution

Mme Michelle Gréaume. L'article L. 141-3 du code de l'éducation dispose que l'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. Par cet amendement, nous proposons d'étendre cette liberté à l'ensemble des établissements publics des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. il est souligné dans l'objet de notre amendement, aujourd'hui, moins de 50 % des élèves du primaire, moins de 20 % des élèves des collèges et moins de 10 % des élèves des lycées participent en Alsace aux cours d'enseignement religieux. En Moselle, cette proportion est identique en primaire, mais inférieure à 10 % au collège ; seuls deux lycées de ce département délivrent encore des cours d'enseignement religieux pour un total de neuf élèves.

C'est d'ailleurs en ce sens que l'Observatoire de la laïcité, en mai 2015, proposait une réforme respectueuse du droit local. Il s'agissait d'inverser la logique, comme nous le proposons dans cet amendement : que les enfants d'Alsace-Moselle souhaitant suivre un enseignement religieux puissent le faire en s'inscrivant dans un cours optionnel. Inscrire dans la loi cette faculté pour tous les établissements serait une mesure de simplification en direction des familles et des équipes pédagogiques. En parallèle, elle s'inscrirait pleinement dans les décisions du Conseil constitutionnel d'avril 2001 et août 2011. Quel est l'avis de la commission de la culture

petite partie de l'explication. Comme vous le savez peut-être, le droit local est constitué de plusieurs strates successives : de textes français qui remontent à Napoléon, puis de textes allemands postérieurs à 1870, puis de textes français après 1918, lorsque l'Alsace est redevenue française, puis de textes allemands de nouveau. Bref, nous sommes face à l'un des éléments du droit local auquel les Alsaciens sont attachés.

J'aime beaucoup la presse, mais j'aimerais bien qu'elle rende compte de la situation telle qu'elle est véritablement, de façon exhaustive. Lorsque, dans une autre question, on demande à ces mêmes Alsaciens s'ils pensent qu'il convient de continuer à

la nature réglementaire de ce dispositif, mais parce que le droit local mériterait une réflexion d'ensemble, comme l'a excellemment rappelé mon collègue alsacien André Reichardt- je ne suis que Lorrain non concordataire ! Cela dit, je voudrais rendre hommage à Mme Assassi et à son groupe, parce que nous avons enfin une explication assez cohérente de l'histoire des strates législatives de ces trois départements d'Alsace et de Moselle. Il y a une solidarité dans le droit local qui interdit de le détricoter par petits bouts ; ce n'est d'ailleurs pas demandé localement. Nous pourrions en revanche- la loi française le permet, notamment par ses dispositifs d'expérimentation -avoir une réflexion d'ensemble sur ce que pourrait être un nouveau droit local. Il appartiendrait évidemment à ces trois départements d'y réfléchir et de faire leurs propres propositions en la matière. Dans l'instant, je vous propose de repousser cet amendement et de consolider le droit local, globalement et en particulier dans son volet

est régi par la loi du 12 février 1873, qui a reçu son ordonnance d'application le 10 juillet 1873, ainsi que par un règlement du 20 juin 1883. L'ordonnance du 10 juillet 1873 dispose, en son article 10 A : « Dans toutes

Mme Jocelyne Guidez. L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation interdit le port de signes religieux ostentatoires dans l'enceinte des établissements scolaires Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. La pratique de la religion étant un sujet particulièrement sensible et intime, il apparaît indispensable de réaffirmer que la logique de médiation, d'explication et de dialogue doit prévaloir dans le cas où un élève contreviendrait à cette interdiction. Il paraît également indispensable d'associer les parents ou les responsables légaux à cette démarche afin que celle-ci soit mieux comprise et donc mieux appliquée. Quel de la culture ? Nous sommes là dans l'application concrète de la loi de 2004, laquelle interdit le port de signes et de tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les collèges et dans les lycées. On peut imaginer que, lorsqu'un élève veut se soustraire à cette interdiction, un dialogue s'établit entre les responsables de l'établissement et les parents. Néanmoins, cela n'est pas inscrit noir sur blanc dans l'article L. 141-5-1, que vous

scolaires. Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont des bénévoles. Ils sont investis d'une fonction officielle : ils veillent aux bonnes conditions de vie de l'enfant, à l'école et autour de l'école, et au respect de la laïcité. Garants des valeurs républicaines, ils agissent en appliquant les principes fondateurs de l'école publique : égalité, gratuité, laïcité. laïcité. Ni usagers, comme les parents, ni directement acteurs, comme les enseignants, ces délégués sont de véritables partenaires de l'école publique et s'associent à la communauté éducative dans le seul objectif de défendre l'intérêt des élèves. Leur indépendance leur donne notamment un rôle de médiateur entre les enseignants, les parents d'élèves, la municipalité et les services académiques. Comme ces délégués sont membres de droit du conseil d'école et membres du conseil départemental de l'éducation nationale, nous proposons qu'ils soient également membres des conseils d'administration des collèges. Nous estimons que leurs compétences concernant les écoles et leur connaissance approfondie du fonctionnement de l'éducation nationale

Monsieur le ministre,

Faut-il pour autant prévoir la systématicité de leur présence dans les conseils d'administration ? Je me pose la question. Vous savez que ma pente est favorable, puisque vous avez rappelé que j'avais

Le projet éducatif territorial permet d'organiser les activités périscolaires, qui ont vocation à s'adresser à tous les enfants. Cet outil, qui rassemble les collectivités locales et la communauté éducative, a pour objectif de favoriser le développement personnel de l'enfant, tant au niveau de ses aptitudes intellectuelles et physiques que de son implication dans la vie en société. Veiller à la qualité des activités proposées fait partie des objectifs du projet éducatif territorial. Par cet amendement, nous souhaitons que figure clairement dans ses objectifs le respect de la charte de la laïcité et du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit ainsi d'appuyer les grandes lignes de ce projet de loi, qui entend notamment réaffirmer les valeurs de la République pour mieux lutter contre les dangers du séparatisme pesant sur certains enfants. Dans cette lutte contre les atteintes à la laïcité, tous les moyens, à tous les niveaux, doivent être mobilisés pour favoriser l'apprentissage précoce du vivre ensemble, garant de la cohésion sociale dans notre pays.

du sens, même si, selon les espaces dans lesquels on se trouve, les règles peuvent être différentes. C'est l'occasion pour moi d'insister sur le fait que

agir sur les facteurs sociaux de la réussite de l'enfant et le faire grandir dans les valeurs de la République. C'est pourquoi agir sur les

de ce concept de laïcité, de ses valeurs et des principes forts qu'il porte, si nous ne sommes pas en mesure de les appliquer dans l'ensemble de la sphère publique ? J'ai notamment à l'esprit le premier rendez-vous

pour rappeler que la laïcité n'est pas à géométrie variable. J'ai même posé la question en tant que président du département, le 2 juin 2015, en préfecture du Pas-de-Calais, en présence du correspondant défense. J'ai demandé simplement que l'on m'indique

avec restauration, j'avais une idée des prix qui pouvaient être pratiqués pour délivrer les repas, et nous étions disposés à ouvrir nos établissements pour accueillir les jeunes. Depuis ce temps-là, chaque année et à chaque session, les jeunes sont accueillis à la maison diocésaine. Je n'ose imaginer, monsieur le ministre, qu'il s'agisse là d'un financement déguisé de la part de l'État

: La parole est à M. Pierre Ouzoulias. L'article L. 912-1-1 du code de l'éducation dispose que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement

Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. » Nous visons les comportements des élèves qui, dans la classe,

De la même façon, nous voyons trop souvent les parents intervenir directement dans la pédagogie de l'enseignant, dans les choix d'oeuvres, dans les disciplines.

une immixtion dans la liberté pédagogique et dans le cours des enseignants tels qu'ils conçoivent de le déployer au cours de l'année. Cet amendement permet de rappeler la liberté pédagogique des enseignants, qui doit être protégée face aux parents et aux élèves. La commission, de manière très cohérente, a émis un avis favorable. Quel est

que le point le plus important se trouve sans doute dans la deuxième phrase, qui impose une obligation de respect vis-à-vis du professeur de la part des élèves, mais aussi de la part de leurs familles. Bien entendu, cette conviction est

terriblement à l'affaire Paty : un professeur exerce sa liberté pédagogique et se trouve contesté par des parents qui s'estiment blessés par le fait que l'enseignant a parlé de liberté d'expression au travers de caricatures.

il s'agit d'une disposition lourde. Nous visons ici quelque chose de plus modeste, qui s'opère directement dans la classe. Il serait complètement aberrant que le texte protège l'enseignant contre son conseil pédagogique

explication de vote. Pour la deuxième fois de la journée, je dis à Pierre Ouzoulias que je regrette de ne pas avoir pensé à écrire la même chose que lui. Je partage totalement son amendement et la manière dont il l'a présenté.

la liberté pédagogique de professeurs qui voulaient conserver des méthodes qui leur appartenaient, pourvu que celles-ci s'inscrivent dans le cadre du respect des programmes et des instructions ministérielles.

des contrôles plus approfondis et plus détaillés. Il me semble donc utile de préciser dans la loi que, lors des contrôles, les missions des inspecteurs de l'éducation nationale doivent être particulièrement orientées vers le respect des principes de la République.

non seulement sur les enjeux de transmission des connaissances, mais aussi sous l'angle du climat scolaire- par exemple, la lutte contre le harcèlement -et du respect des valeurs de la République et de la laïcité.

La laïcité est un principe qui découle de la liberté. Si nous faisons cette erreur d'appréciation, ce n'est pas la peine de discuter comme nous le faisons depuis des jours.

aux grandes questions sociétales et, surtout, de les problématiser pour qu'ils puissent les comprendre et les assimiler.

Ces enfants et adolescents laissés libres de leurs mouvements ne suivent plus régulièrement leur scolarité et se livrent à des troubles à l'ordre public pouvant aller jusqu'à entraîner la mort. Dans ce contexte, les parents doivent être convoqués par l'inspecteur d'académie, qui aura ainsi la possibilité d'apprécier si les parents sont dépassés par leur enfant ou s'ils n'ont pas l'intention d'assumer leurs responsabilités parentales. L'article 227-17 du code pénal dispose que « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire [ ...] à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil Cet amendement a pour objet de donner un outil supplémentaire à l'inspecteur d'académie, à savoir la possibilité de demander la suspension totale ou partielle des prestations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire, s'il est clairement démontré que les parents ne remplissent plus leur rôle d'éducation et de soins. Je souligne bien qu'il s'agit d'une possibilité, et non d'une mesure automatique. Bien entendu, les parents en difficulté, essentiellement les familles monoparentales, pourront être aidés s'ils manifestent la volonté d'essayer de rétablir la situation. Les dispositifs existants le permettent. En revanche, en cas de démission parentale, il n'y a aucune raison de leur apporter une aide qui, de toute évidence, ne va pas à l'éducation de l'enfant. Les prestations qu'ils perçoivent au titre de cet enfant pourront donc être diminuées, voire supprimées.

l'objectif de cet amendement est de lutter contre l'absentéisme, celui des allocations familiales n'est pas de faciliter le présentéisme.

on ne vit pas des allocations familiales ; on ne fait pas des enfants pour s'enrichir grâce aux allocations familiales ! La volonté de lutter

autant, la suppression des allocations familiales répond-elle à cette impérieuse nécessité de lutter contre l'absentéisme, le décrochage scolaire, voire le retrait de l'école par un certain nombre de familles ?

une famille où les parents n'arrivent pas à obtenir de lui qu'il se rende quotidiennement à l'école. Je ne crois pas qu'il y ait des parents indifférents au fait que leur enfant n'aille pas à l'école. Je ne crois pas qu'il y ait des parents laxistes ou complices.

Nous visons tous ensemble le même but : protéger les enfants contre la déscolarisation et contre les familles qui n'ont pas l'autorité suffisante. Mais ce n'est pas en supprimant une ressource qui n'est pas liée

Je crois revivre le débat que nous avons eu dans cet hémicycle quand j'ai eu l'honneur de présenter le dispositif du contrat de responsabilité parentale en 2006.

à suspendre les allocations familiales des parents : sur les 6 280 seconds signalements adressés aux inspecteurs d'académie, 147 demandes de suspension 51 ont été effectives. Vous voyez bien que le coeur du dispositif n'est pas la sanction. Il s'agit précisément d'éviter la sanction, qui n'est prévue qu'en dernier recours. Très bien ! Le coeur du dispositif, c'est le contrat de responsabilité parentale. Il s'agit d'accompagner les parents pour qu'ils se ressaisissent, de les aider

l'inspiration de cet amendement est parfaitement humaniste. Oh ! Nous devrions l'admettre sur toutes les travées au lieu de réactiver les vieux réflexes gauche-droite d'antan. Il s'agit simplement de trouver la bonne mesure pour faire face à l'absentéisme.

De plus, ce n'est pas une suppression, mais une aide éducative qui est engagée sans préjudice de toutes les autres mesures qui doivent être prises en matière de signalement et de prévention.

la reconnaissance par la Nation de l'investissement éducatif des parents à l'endroit de leurs enfants qui feront les adultes de demain. Je considère qu'il est tout à fait logique que les allocations familiales servent le but pour lequel elles ont été créées, c'est-à-dire aider les familles sur le plan pécuniaire, mais aussi marquer un acte de reconnaissance de la Nation envers ces éducateurs que sont les parents.

en tant qu'ancien ministre de la ville, de mes nombreuses visites dans les quartiers Nord de votre ville. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler dans quel état se trouvaient les écoles publiques de ces quartiers. Ça n'a

de vote. Chers collègues, je souhaite vous poser une question : croyez-vous qu'on peut éduquer des parents en les punissant ? Oui ! Nous avons pourtant voté des textes anti-punitifs concernant les enfants.

nous poussons encore plus dans la détresse, aussi bien alimentaire que psychologique, des parents qui n'arrivent pas à gérer l'assiduité de leurs enfants à l'école.

entre les autorités académiques, celles du département et celles des allocations familiales. Pourquoi ne faites-vous pas confiance à tous les acteurs de ce système, qui disposeront d'une procédure